des papiers graphiques n'est que de 62 %. Ce faible taux de performance peut-il être amélioré en faisant contribuer financièrement le secteur de la presse à la gestion des déchets ? Je ne le pense pas.

La révision de la directive européenne sur les déchets, intervenue en 2018, qui a imposé le caractère financier des écocontributions, a conduit les pouvoirs publics à questionner ce modèle.

La présente proposition de loi, ainsi qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale, prévoyait d'extraire les publications de presse de la REP papier, en contrepartie de la conclusion d'une convention de partenariat avec l'État afin de déterminer les conditions de la mise à disposition des encarts publicitaires ainsi que des critères de performance environnementale. La commission l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a souhaité pour sa part maintenir les publications de presse dans la REP et introduire une modulation des contributions sous la forme d'une prime accordée notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts d'information et le respect de critères de performance environnementale. Cela inquiète à double titre : la presse ne dispose plus de la garantie de pouvoir contribuer en nature et les autres producteurs de la filière devraient contribuer à sa place. Il s'agit de la mutualisation des coûts introduite en commission. Nous viendrions ainsi fragiliser le secteur de la presse alors qu'il vient déjà de subir le doublement du prix de la tonne de papier en l'espace d'une année dans un contexte de hausse du coût de l'énergie. Nous proposerons donc de rétablir la rédaction de l'article 1 retenue par l'Assemblée nationale, qui nous semble constituer le meilleur compromis. En aucun cas, cela ne doit être perçu comme un blanc-seing puisque les critères de performance environnementale continueront de s'appliquer. D'aucuns évoquent un « dangereux précédent » pour les autres filières. Mais c'est à nous, en tant que législateur, de ne pas céder le moment venu à des dérogations qui ne seraient pas justifiées. Pour ce qui est de la presse, nous sommes convaincus de l'inadaptation de l'écocontribution financière. Peut-on considérer les éditeurs de presse comme des pollueurs et les journaux comme de simples déchets ? Je ne le pense pas Si l'on veut améliorer nos performances de collecte du papier, commençons par assurer la collecte séparée de ce flux, comme cela se fait dans d'autres pays européens. Appliquons les amendes prévues par le droit en vigueur lorsque le tri n'est pas réalisé. Mes chers collègues, les « taxes », entendues au sens large, ne peuvent à elles seules résoudre tous les problèmes. J'en viens au deuxième sujet soulevé par la proposition de loi : la fusion des filières emballages ménagers et papier pour des raisons administratives et pour favoriser les synergies. Une étude d'impact aurait été appréciable. Pour cela, le dépôt d'un projet de loi, de préférence avant la fin du dispositif dérogatoire qui avait été adopté dans la loi Agec, n'aurait pas été superflu. Cela nous aurait évité d'adopter une loi rétroactive alors que le Gouvernement disposait de trois ans pour se pencher sur la question. Nous avons été alertés sur les risques de la fusion financière de ces deux filières. En effet, cela pose des problèmes d'équité : chaque filière doit couvrir les coûts dont elle est responsable. Pour conclure, dans un contexte de déclin continu des ventes de journaux traditionnels au profit des réseaux sociaux et des, ne sacrifions pas la presse pour une plus-value plus qu'incertaine Attaché au rôle démocratique de la presse, qui informe nos concitoyens et les accompagne dans l'exercice de leur souveraineté, le groupe du RDSE déterminera sa position en fonction de l'issue des débats.

nous débattons aujourd'hui de la proposition de loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier. Je tiens tout d'abord à saluer l'excellent travail de notre rapporteure, Marta de Cidrac, qui a su avec force et détermination mener ce travail législatif,

Ce principe est fondamental dans le droit de l'environnement. Il est devenu l'un des quatre grands principes généraux du droit environnemental avec la loi Barnier de 1995 et est consacré dans l'article 4 de la Charte de l'environnement qui dispose : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi. » Ce texte permet également la fusion des filières REP, qui doit être source de simplification et de synergie des acteurs, afin d'améliorer la chaîne du recyclage et de permettre l'efficacité environnementale. Ensuite, ce texte prévoit d'aider le secteur de la presse, tout en le maintenant dans la REP, la modulation des contributions financières de la filière REP pour les produits contribuant à une information d'intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets. Cela passe notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts, sous réserve de respecter des critères de performance environnementale fixés par décret. Ce dispositif protège alors le secteur de la presse, qui fait aujourd'hui face à des difficultés conjoncturelles et structurelles, comme de nombreux autres secteurs d'activité, tout en le conservant dans le dispositif REP : nul ne peut s'en exonérer ou s'en extraire. Enfin, cette proposition de loi garantit le financement et le service public de gestion des déchets (SPGD) géré par les collectivités territoriales.

En effet, la directive européenne qui nous conduit à étudier ce texte était connue depuis longtemps et nous attendions de la part de l'État plus d'anticipation pour répondre à cette problématique. En tout état de cause, grâce au travail de notre rapporteure, Marta de Cidrac, ce texte préserve l'intégrité de la REP en réintégrant la presse en son sein. Il est financièrement neutre pour le service public de gestion des déchets et offre des garanties environnementales, en conditionnant l'octroi des primes. Pour toutes les raisons que j'ai invoquées, le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi, amendée par notre commission, portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier.

Il est prouvé que l'activité humaine a un rôle important dans ce dérèglement. Je rappelle que le plus grand des pollueurs reste la Chine, qui représente à elle seule 33 % des émissions mondiales de CO2 soit 12 milliards de tonnes,

et l'ensemble de la biodiversité. Nous subissons déjà un manque inquiétant d'eau alors que commence à peine le printemps. Certains territoires sont déjà en restriction. Cela menace notre souveraineté alimentaire et plus largement notre économie.

existent pour cela -à une ressource en eau moins abondante. En effet, c'est bien d'adaptation qu'il est question. Nous devons faire évoluer nos modes de vie, nos industries, et cela passe par une économie circulaire.

J'en profite pour saluer le travail de la rapporteure et de la commission. Le texte a été totalement réécrit afin de trouver un équilibre différent tout en gardant l'objectif principal de la fusion. En ce qui concerne l'exonération de la presse- le point du texte qui a suscité le plus de discussions -, beaucoup étaient d'accord pour dire qu'une exclusion totale n'était pas la solution, en mentionnant le risque de fragilisation du système et de création d'un précédent qui en entraînerait inévitablement qui en entraînerait inévitablement d'autres. Mais nous connaissons les difficultés du secteur de la presse écrite, et nous devons les prendre en considération. L'importance de la presse dans un pays et dans une démocratie est capitale. L'information est la clé d'un citoyen éclairé ; celle du public sur la prévention et la gestion des déchets en fait bien sûr partie, et nous aurions souhaité le rétablissement de l'article 1. Mes chers collègues, nous sommes tous concernés par la gestion de nos déchets,

équilibre entre, d'une part, le principe pollueur-payeur, qui doit assurer au service public de gestion des déchets une juste contribution financière des producteurs et des metteurs sur le marché à la prise en charge des déchets résultant de leurs produits, et, d'autre part, la nécessaire sauvegarde de la presse écrite, qui est en forte difficulté. Le journal, puisqu'il est essentiel à la vie libre des idées, à la culture et à la vitalité démocratique, n'est ni un produit comme un autre- cela a été dit -ni un déchet comme les autres. Cet équilibre nécessite, à la fois, de ne pas aggraver fortement les difficultés engendrées par la crise majeure de la presse, et particulièrement de la presse régionale, et de répondre aux besoins du service public de gestion des déchets, assuré par les collectivités territoriales pour réduire, collecter, trier et recycler, les collectivités ont besoin de contributions financières, de ressources à la hauteur. En France, l'organisation de la prévention et de la gestion des déchets repose intégralement sur le mécanisme des filières REP, qui est né dans les années 1990, qui, ayant fait ses preuves, a ensuite été généralisé en Europe par la directive sur les déchets. Ces derniers jours, on a pu mesurer dans les rues de Paris la quantité astronomique de déchets accumulés en très peu de temps. Il est indispensable que les producteurs intègrent un coût de prévention et de gestion des déchets : ils doivent être incités à concevoir des produits moins générateurs de déchets, triables, recyclables, réemployables. En excluant la presse de la REP, le texte dans la version de l'Assemblée nationale créait non seulement un recul environnemental, mais également un précédent risqué, qui risquait de déstabiliser les REP et d'entraîner un manque à gagner bien lourd pour les collectivités. Cela serait la première fois qu'un gisement serait retiré de la REP, ouvrant la porte à des exemptions et à des exonérations d'autres secteurs, au détriment de l'environnement et des collectivités.

La proposition de l'Assemblée nationale en la matière n'était acceptable ni du point de vue des collectivités, qui resteraient privées d'une part des contributions financières, ni du point de vue de l'intérêt général, encadré par la loi Agec et la directive sur les Il s'agissait d'une astuce qui déresponsabilisait, en tout cas financièrement, des producteurs de déchets. Pour autant, nul ne peut ignorer les difficultés de la presse. En dix ans, les cours du papier se sont envolés, les ventes et le lectorat se sont réduits : au total, le nombre d'exemplaires imprimés a diminué de 41 %. Le tour de passe-passe proposé par Mme la rapporteure, est plus juste, et donc plus judicieux, puisqu'il ne se ferait pas sur le dos du service public de gestion des déchets. La presse écrite s'en sortirait sans dommage, car ses contributions financières pourraient être écomodulées, notamment par des encarts gratuits d'information et de sensibilisation citoyenne sur la prévention et la gestion des déchets. Les primes ainsi consenties seraient compensées par une augmentation des contributions des autres metteurs sur le marché soumis à la même filière REP, par le renforcement des pénalités de pratiques polluantes ou par une augmentation de la contribution de base.

D'abord, sur la question de la fusion des deux filières emballages et papier. Cette fusion prend tout son sens avec le mécanisme proposé, les contributions financières au sein d'une filière étant basées sur un principe de solidarité globale entre les acteurs. Néanmoins, il faut le dire, certains acteurs de la filière papier sont inquiets. Les deux types de déchets ont leurs spécificités de tri et de traitement. Il est peut-être important de maintenir des critères d'agrément distincts pour contrôler le respect des obligations.

Autre interrogation : celle du taux de couverture. La loi fixe le taux de couverture des coûts de gestion des déchets supportés par les collectivités à 50 % pour les papiers et à 80 % pour les emballages. À ce jour, ce taux n'est pas respecté par les éco-organismes : il est d'environ 20 % pour les papiers et de 50 % pour les emballages. L'État ne joue pas son rôle de régulateur. Là se joue notre service public de gestion des déchets.

déposés sur la proposition de loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier et amplification des encarts publicitaires destinés à informer le public sur la transition écologique. Le texte Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoit le regroupement des deux filières, aujourd'hui distinctes, dans un triple but. D'abord, apporter une simplification administrative aux collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets : elles n'auraient plus à contractualiser qu'avec un seul éco-organisme. Puis, faire suite à la loi Agec, qui est venue harmoniser les systèmes de collecte des déchets pour les deux éco-organismes sur l'ensemble du territoire. Enfin, mutualiser les coûts, alors que le remplacement des emballages plastiques se fera par un recours accru aux papiers et cartons. Notre groupe se prononce en faveur de cette unification des deux REP, soutenant l'opportunité de la synergie ainsi recherchée. La proposition de loi entend par ailleurs exonérer le secteur de la presse du paiement de la contribution financière, ce dernier en étant redevable depuis le début de l'année, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Pour ce faire, elle vient substituer à l'application du principe pollueur-payeur aux publications de presse- en vigueur depuis le 1 janvier 2023, -une obligation de mise à disposition gratuite par la presse d'encarts publicitaires visant à informer les lecteurs sur des problématiques environnementales. Concrètement, la proposition de loi tend à exempter la presse de la filière REP des papiers graphiques, à la condition qu'une convention de partenariat soit signée avec l'État. Cette convention devrait engager la presse à mettre à disposition gratuitement des encarts sur le tri des déchets, l'économie circulaire et la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité, au bénéfice des collectivités territoriales- notamment des intercommunalités -et de la communication des filières REP et des associations agréées pour la protection de l'environnement. Ce partenariat permettrait de définir, dans le même temps, des critères de performance environnementale que les publications s'engageraient à respecter. Il s'agira de maintenir les obligations de transformation industrielle du secteur en matière de taux de recyclage et de limitation des perturbateurs du recyclage. Ce serait dans les faits une continuation du système actuel de la contribution en nature, mais portée différemment, avec l'objectif de donner à la presse les outils pour prendre pleinement part aux défis de la transition écologique. Pourquoi une telle prorogation ? En raison du contexte, constaté par tous, très dégradé de ce secteur crucial.

La loi Agec de 2020, en anticipant sur l'application du droit européen, a cependant mis un terme à ce régime spécifique en prévoyant qu'à compter de cette année l'écocontribution de la presse devait être numéraire. Nous y sommes, et c'est pourquoi une nouvelle réponse doit être proposée. La presse écrite, nationale et régionale, est un pilier de notre démocratie ; elle est aussi financièrement exsangue. Au sein de notre commission, madame la rapporteure, vous avez défendu le nécessaire soutien et à la presse et aux collectivités territoriales, qui se trouveraient privées d'une nouvelle ressource. Rappelons ici que, pour les raisons invoquées précédemment, il s'agit pour les collectivités non pas d'une perte de revenus, mais d'un manque à gagner. Celui-ci représente 0,25 % du coût total du service de gestion des déchets. Vous avez par conséquent prévu, tout en maintenant la presse dans la REP nouvellement créée afin d'éviter un « précédent d'exonération », une modulation sous forme de prime du montant de la contribution financière des produits assujettis.

Tout d'abord, cet équilibre pourrait contrevenir à la directive européenne sur les déchets de 2018, ce qui entraînerait un risque important de contentieux juridique. Si le code de l'environnement prévoit le possible recours à une modulation de l'écocontribution, celle-ci doit être effectuée « en fonction de critères de performance environnementale liés au produit en question, sans que des actions de communication ou de sensibilisation aux consommateurs soient expressément prévues. En cas de recours, la presse se retrouverait à devoir payer une écocontribution de façon rétroactive, sans solution de remplacement. Ensuite, selon les critères établis, le bonus pourrait bénéficier à d'autres organismes que celui de la presse, ouvrant là aussi un précédent, mais cette fois-ci au sein même de la REP nouvellement constituée. Ce risque d'appel d'air aurait des conséquences sur le montant global des écocontributions, ce qui contreviendrait aux objectifs environnementaux. Enfin, il incomberait aux autres opérateurs d'être solidaires du secteur, alors que certains d'entre eux sont soumis à des contraintes économiques importantes. Au regard de ces observations, notre groupe votera majoritairement contre ce dispositif. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la loi Agec a refondé certains principes de l'économie circulaire, tout en renforçant la responsabilité des metteurs sur le marché dans la gestion des déchets, de la création du produit à sa fin de vie. En réaffirmant haut et fort le principe du pollueur-payeur, le Sénat s'est inscrit dans les enjeux de notre siècle, soucieux de l'impact environnemental de la production de biens. Cependant, bon nombre de filières REP peinent encore à voir peinent encore à voir le jour en dépit de l'entrée en vigueur de celles-ci au 1 janvier 2023. Je pense par exemple à la REP bâtiment, à la REP jeux et jouets ou encore à la REP textile. Autre dispositif imposé par la loi Agec qui nous intéresse ici : la fin du régime dérogatoire ouvert à la presse en 2015, qui lui permettait de contribuer sous la forme de prestations en nature et non par le versement d'une écocontribution. Ainsi, en l'état du droit, depuis le 1janvier 2023, le versement de l'écocontribution doit obligatoirement avoir un caractère financier pour la presse écrite. C'est le point nodal de cette proposition de loi, qui vise à exempter la presse de cette écocontribution par la réintroduction d'un régime dérogatoire en raison des difficultés économiques rencontrées par ce secteur d'activité. Il s'agit de permettre à un secteur de déroger à un principe encore jeune et imparfaitement appliqué par les industriels. Acter cette exemption crée un précédent fâcheux, qui, mécaniquement, suscitera d'autres demandes émanant de secteurs fragiles au sein d'autres REP, voire d'acteurs issus de la REP papier, comme l'industrie papetière, qui traverse une importante crise en continuant malgré tout à payer son écocontribution.

un impact financier sur les collectivités territoriales chargées de la collecte, du tri et du recyclage des papiers par le biais du bac jaune. Défenseurs du service public des déchets, nous souhaitons profiter de ce débat pour mettre l'État devant ses responsabilités. Exempter purement et simplement la presse écrite ou tout autre acteur n'est pas une solution pérenne, car cela fragilise à court terme nos filières REP. Si le Gouvernement estime que les spécificités du secteur de la presse écrite justifient une telle exemption au principe général du pollueur-payeur, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il doit prendre en charge le coût de cette décision et, en aucun cas, ne doit la faire peser sur les autres contributeurs de la future REP fusionnée. Deuxième point dur de ce texte : la fusion des deux REP papier et emballages ménagers. Cette mutualisation des filières n'est pas demandée par les acteurs concernés. Je demeure dubitatif quant à cette simplification effectuée sans concertation, sachant que les deux cahiers des charges sont d'ores et déjà en vigueur, qu'ils sont utiles aux acteurs et qu'ils coexisteraient dans une filière unifiée. Ainsi, nous tenterons lors du débat de préserver la distinction entre les deux flux financiers, supprimée par la rapporteure, afin de prendre en compte les spécificités de ces deux filières, ainsi que la différence importante de leurs poids financiers, allant du simple au décuple. Nous pouvons tout de même saluer les efforts de la rapporteure Marta de Cidrac qui, lors des travaux de notre commission, a démontré sa volonté de trouver un consensus acceptable par l'ensemble des parties, même si des zones d'ombre persistent.

a choisi de confier à l'éco-organisme le soin d'accorder ou non ces primes en fonction du futur cadre fixé dans le décret. Mais mon inquiétude vis-à-vis de cette nouvelle écriture réside dans la porte laissée ouverte à l'ensemble des metteurs sur le marché de la filière REP, et pas seulement à la presse écrite.

entre l'éco-organisme agréé, les collectivités territoriales et les entreprises concernées, afin de permettre au secteur de la presse de payer son écocontribution pour tout ou partie en nature, sous la forme d'encarts publicitaires visant à favoriser les écogestes et le recyclage. S'il faut protéger le secteur de la presse, qui traverse bel et bien une crise difficile, assurons-nous, mes chers collègues, de bien circonscrire cette exemption pour garantir le respect du principe du pollueur-payeur qui nous rassemble et pour rester en conformité avec la loi Agec Cette précision permettra de marquer notre volonté commune de ménager, à la fois, la presse écrite et le service public de gestion des déchets, auquel nous sommes tous très attachés sur ces travées. En raison des éléments que je viens d'indiquer, notre groupe s'abstiendra sur ce texte.

Je le dis pour souligner le fait que, parmi toutes les urgences en cours, et pour lutter contre le dérèglement climatique, très corrélé à notre utilisation des ressources naturelles, nous utilisons le temps parlementaire sous un angle qui peut paraître légèrement décalé, même si personne ne remet en cause ici la fusion des filières. Il faut, c'est vrai, souligner l'utilité de faire contribuer les producteurs de déchets plutôt que les consommateurs, qui n'ont parfois pas d'autres solutions que de consommer des produits emballés, voire suremballés.

Alors, fusionner les filières, pourquoi pas ? Il y a sans doute un enjeu de lisibilité, d'efficacité et d'économie sur les coûts de fonctionnement qui pose une vraie question : comment financer la collecte des déchets si ces deniers diminuent ? Un rapport de la Cour des comptes de septembre dernier pointe cet enjeu et rappelle également un argument de bon sens : le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas.

Dans de nombreuses intercommunalités, le ramassage des déchets se fait plus rare, faute de moyens ; cette dégradation et le surcoût du service sont supportés par les usagers.

mérite qu'on le questionne. C'est ce qu'avait fait l'Assemblée nationale, dont le travail a été reconsidéré ici pour préconiser des dispositions qui demeurent floues-

Une vraie réforme doit être menée sur le sujet, mais la discussion ne peut avoir lieu uniquement sur la question de l'écocontribution ou de l'écomodulation.

la présente proposition de loi, qui est en réalité un texte voulu par le Gouvernement, a deux objets d'inégale importance. Le premier de ces objets est la fusion de deux filières à responsabilité élargie du producteur, les REP d'emballages ménagers et de papier. Cette fusion est rendue souhaitable par l'harmonisation des modalités de collecte de ces deux types de déchets à l'échelle nationale depuis le 1 janvier 2023. Ainsi, cette simplification administrative devrait faciliter la tâche des collectivités, qui pourront contractualiser avec un éco-organisme unique, un contrat unique. Elle contribuera plus globalement à l'harmonisation de la collecte des déchets d'emballages et de papier sur l'ensemble du territoire national. Cela a déjà été dit, mais je tiens tout de même à souligner que cette fusion intervient à un moment stratégique pour les filières concernées celui de la mise en place envisagée de la consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques, qui ne concernera pas, par définition, la filière des papiers graphiques ; et celui de l'expérimentation du « Oui pub », institué par la loi Climat et résilience, qui doit aboutir à la fin de 2024 et qui, elle, ne concernera pas la filière emballages ménagers. Madame la secrétaire d'État, nous comptons sur votre vigilance pour que, dans ce contexte, la fusion ne perturbe pas le fonctionnement des filières. J'en viens au second enjeu de la présente proposition de loi, à nos yeux le plus stratégique, celui qui concerne spécifiquement le secteur de la presse. Jusqu'au 1 janvier dernier, les éditeurs de presse étaient exemptés d'écocontribution. Plus précisément, il leur était possible de s'en acquitter en nature, par la mise à disposition d'encarts publicitaires relatifs aux bons gestes de tri. Mais la loi du 10 février 2020, transposant la directive Déchets de 2018, a mis un terme à ce régime dérogatoire en disposant qu'à partir du 1 janvier 2023, l'écocontribution versée par les éditeurs de presse devrait obligatoirement avoir un caractère financier. Or chacun a bien conscience aujourd'hui que la presse écrite est en grande difficulté- tous les orateurs l'ont signalé. Je veux parler des difficultés structurelles liées à la fonte tendancielle du lectorat, du lectorat, aujourd'hui aggravées par l'impact de chocs conjoncturels que sont le quasi-doublement du prix du papier et l'envolée des prix de l'énergie. Compte tenu de cette situation et de l'importance que revêt la presse, particulièrement dans nos territoires ruraux, il nous faut continuer de soutenir le secteur en l'exonérant d'écocontribution. Cela ne fait pas débat. Ce qui est moins consensuel, c'est de savoir comment ! La proposition du Gouvernement n'était pas acceptable pour les représentants des collectivités que nous sommes. En effet, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale sortait le secteur de la presse de toute REP pour continuer de l'exonérer sans être en contradiction avec la directive européenne. Résultat : avec ce dispositif, c'est aux collectivités locales de payer puisque, évidemment, l'État ne propose aucune compensation. C'est pourquoi nous soutenons vivement la solution proposée par notre rapporteure, dont je salue au passage la qualité du travail. Elle prévoit d'intégrer pleinement la presse écrite dans la nouvelle REP fusionnée et de moduler son écocontribution en contrepartie d'encarts d'information sur le recyclage. Cette solution est un qui ménage tous les intérêts : celui de la presse et des collectivités, bien sûr, mais aussi celui de l'environnement, car sortir la presse de sa REP créerait, nous le savons tous, un dangereux précédent. Ce serait ouvrir une brèche dans toute la politique du recyclage. Demain, tout secteur en difficulté pourrait légitimement se prévaloir de la jurisprudence « presse papier » en échange d'encarts sur son.

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier. Je tiens à saluer le travail remarquable de notre collègue Marta de Cidrac, qui a su trouver un subtil équilibre entre la nécessité, pour la France, de se conformer au droit européen, de préserver la situation, au demeurant très fragile, des éditeurs de presse et de protéger le service public de gestion des déchets, géré par les collectivités territoriales. Le compromis auquel notre rapporteure est parvenue pour concilier ces enjeux en apparence contradictoires permet de protéger la presse sans l'exonérer pour autant des responsabilités qui lui incombent en tant que producteur de déchets. Je précise que les collectivités territoriales, dont le Sénat est le représentant attentif, ne perdront rien à l'occasion de la mise en oeuvre de cette réforme. Le manque à gagner lié au versement des primes, estimé entre 22 et 26 millions d'euros, sera en effet mutualisé entre l'ensemble des metteurs sur le marché relevant de cette nouvelle filière. La proposition de loi de nos collègues députés était juridiquement contestable. Elle maintenait la presse dans un statut dérogatoire, permettant aux éditeurs de s'acquitter d'une prestation en nature, sous réserve qu'ils signent avec l'État une convention de partenariat prévoyant la mise à disposition gratuite

au 1 janvier 2023, la possibilité de contribuer en nature étant en contradiction avec la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Le dispositif retenu par notre rapporteure prévoit que les publications de presse seront effectivement soumises aux obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs et, en particulier, à une contribution financière versée à un éco-organisme. Toutefois, le montant de cette contribution pourra être modulé, la modulation prenant la forme d'une prime accordée par l'éco-organisme, dès lors que les produits relevant de la nouvelle REP fusionnée contribueront à une information du public d'intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets. Les tarifs appliqués aux éditeurs de presse tiendront compte également des performances environnementales de leurs produits, l'objectif étant, bien entendu, de favoriser les produits vertueux au détriment des produits difficiles à recycler. Les critères de l'écomodulation devraient porter sur l'origine des matériaux utilisés lors de la conception, la recyclabilité des produits et la présence, après recyclage, de substances susceptibles de compromettre l'utilisation du matériau recyclé. Nous l'aurons compris, la modulation vise tout autant à favoriser l'écoconception des produits qu'à améliorer leur réemploi ou leur recyclabilité. Les livres, traditionnellement exemptés en raison de la fragilité économique du secteur, sont maintenus hors du champ de la filière REP. Je m'en réjouis à titre personnel : l'édition fait face à des difficultés conjoncturelles importantes, comme la forte hausse du prix du papier et des coûts d'impression ; elle ne résisterait pas à de nouvelles contraintes financières. En outre, cette exemption me semble aller de soi, le livre étant un produit durable qui se retrouve rarement dans les conteneurs de collecte. Avec les améliorations apportées par Mme de Cidrac au texte initial, c'est tout le secteur de la presse papier, économiquement mis à l'épreuve depuis plusieurs années en raison de l'évolution des usages de lecture et de la concurrence des plateformes numériques, N'oublions pas, mes chers collègues, ce que la vitalité de notre démocratie doit à la presse. La liberté de cette dernière, son pluralisme et son indépendance sont garantis par notre Constitution. Il nous fallait trouver une solution respectueuse de nos engagements européens, soucieuse de l'avenir de la presse et protectrice du service public de gestion des déchets géré par les collectivités territoriales. Elle est présente dans le texte amendé par la commission. En conséquence, je lui accorde sans réserve mon soutien. La parole

allant des microplastiques, présents aussi bien dans les eaux de l'Arctique que dans les glaces au sommet de l'Everest, aux poubelles que nous enfouissons encore massivement dans nos territoires. La grève des éboueurs a le mérite de nous montrer ce que nous ne voulons pas voir, à quoi nous ne pensons pas, à savoir cette quantité de déchets qui est le résultat de notre surconsommation et du tout-jetable. Ce n'est tout simplement plus supportable. Le maître mot reste d'abord, encore et toujours, de les réduire. Il est urgent que tout le monde raisonne de cycle de vie. Il faut que chacun assume sa part dans la gestion des déchets, aussi bien les metteurs sur le marché que les consommateurs, auxquels- il est vrai -on impose trop souvent certains modes de consommation générateurs de rebuts. Chacun doit être responsable. Ce principe est celui du pollueur-payeur, acté dans la loi Agec.

peinent à se mettre en place. On est donc très loin du compte. Tout le monde est en retard. De plus, pour les collectivités qui gèrent la collecte des déchets, tout se complexifie avec l'explosion des coûts, notamment de l'énergie, avec la TGAP qui s'envole et un marché des matières fluctuant et instable. L'équation est très difficile à résoudre

La dissymétrie de volume et de valeur est grande : même si la presse ne représente que 20 % de la REP papier, est-il concevable de sortir un gisement de la filière alors que nous sommes en train de bâtir un dispositif qui englobe l'entièreté du cycle de vie de ce que nous produisons ? Est-ce que la notion même d'économie circulaire, pensée dans sa globalité, n'est pas en quelque sorte remise en cause ?

que nous entrons dans le dur face aux enjeux actuels d'écologie, d'économie et de démocratie. Effectivement, les titres de presse engagés, militants et originaux qui font vivre notre démocratie en donnant d'autres points de vue sur le monde sont diffusés en petit nombre. Cette richesse doit être protégée, cultivée et garantie. Comme le rappelle la Cour européenne des droits de l'homme, ce pluralisme est l'un des éléments constitutifs de la démocratie. Que l'État prenne ses responsabilités ! Cela dit, la compensation en nature par des encarts publicitaires, qui donne lieu à la réduction de l'écocontribution de la presse, représente un manque à gagner pour les collectivités. Ce n'est pas un petit sujet.

dont le journal s'exonère. En l'état, ces encarts ont-ils réellement un effet positif ? Leur contenu ne devrait-il pas être un tant soit peu contrôlé pourquoi pas, inspiré des rapports du Giec, dont le dernier a été rendu public hier ? Le monde dans lequel nous vivons, celui du réchauffement climatique, de l'accumulation des déchets, de trop nombreuses pollutions diffuses et insidieuses, et de la diminution des ressources nous oblige. Le cap ambitieux et vertueux des « trois R »- réduction, réemploi, recyclage recyclage -doit absolument être maintenu en respectant scrupuleusement l'ordre de priorité. Alors que nous entamons un chemin qui se veut plus vertueux, réaliste et responsable, mais qui demeure

L'examen de cette proposition de loi issue de l'Assemblée nationale ne peut, sur le principe, que me satisfaire pleinement puisqu'elle reprend la recommandation n° 6 du rapport d'information, que j'ai présenté devant la commission de la culture et qui a été adopté à l'unanimité le 20 juillet dernier. Quel était le sens de cette recommandation ? Je rappellerai quelques évidences, que je suis- hélas ! -conduit à marteler bien trop régulièrement. La presse n'allait déjà pas très bien ces dernières années, avec des recettes divisées par huit depuis 2000 elle est désormais dans une position dramatique du fait des conséquences de l'inflation qui sont venues percuter de plein fouet le coeur de son modèle économique. En effet, avec l'explosion des prix du papier, des titres strictement à l'équilibre financier plongent désormais dans le rouge ; les autres reportent des investissements pourtant nécessaires. Fort de ce constat, hélas ! toujours plus d'actualité, j'ai proposé plusieurs mesures d'accompagnement. Je réfute, par ailleurs et par avance, tout procès en dépenses excessives. De fait, la presse aurait dû bénéficier d'un crédit d'impôt de 150 millions d'euros, qui a été presque sciemment complexifié avant d'être, finalement, annulé. Je veux également mentionner les 500 millions d'euros d'amende infligés par l'Autorité de la concurrence en juillet 2021 à Google pour non-respect d'injonctions au titre de la rémunération des droits voisins la presse n'a jamais autant rapporté au budget de l'État ! Dans ce contexte, il a paru à la commission de la culture que la fin, au 1 janvier 2023, du régime de compensation de l'écocontribution en nature à Citeo à Citeo tombait plus que mal, et qu'il convenait de s'assurer que la presse ne soit pas frappée d'une nouvelle taxe d'une vingtaine de millions d'euros. Notre collègue Marta de Cidrac a mené- je dois le reconnaître -un remarquable travail, tant juridique que politique, et je loue sa compréhension des enjeux relatifs non seulement à l'écologie, mais également à la presse. En effet, elle s'est trouvée face à une équation cruelle : une fois admis que la presse ne devait pas payer, sur qui doit retomber la charge ? Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, le payeur est la collectivité locale, qui a engagé de lourdes dépenses pour assurer la collecte et le recyclage des déchets et qui ne recevrait donc pas les sommes prévues. cette chambre les représentants des élus locaux et les défenseurs d'une décentralisation souvent piétinée par des gouvernements toujours prêts à mener des politiques d'autant plus ambitieuses qu'elles se font aux frais du contribuable local. Dès lors, je comprends l'émotion suscitée par le texte de l'Assemblée

l'organisation de la fusion des filières REP papier, comprenant les producteurs de papier graphique, et REP emballages ménagers, d'autre part, un soutien indirect au secteur de la presse en prolongeant pour celui-ci la possibilité de payer son écocontribution non en numéraire, mais en nature, par la mise à disposition gratuite d'encarts publicitaires faisant la promotion de la transition écologique.

Il n'y aurait désormais plus qu'une seule filière pour un seul bac jaune puisque tous les papiers graphiques et les emballages en carton ou en papier seraient collectés, triés et recyclés de manière commune. Naturellement, ce dispositif de fusion peut paraître séduisant sur le papier. Pourtant, il n'a été réclamé par aucun acteur de l'une des deux filières, ni par les éco-organismes, ni par les collectivités, ni même par l'industrie papetière. Il a aussi été critiqué par de nombreuses associations d'élus qui considèrent qu'il représente une atteinte, voire une menace à la mise en place par les collectivités de la filière REP. Cette crainte porte sur une nouvelle hausse des coûts supportés par les collectivités et sur un manque de contrôle du respect des objectifs environnementaux de ces filières. En effet, la fusion risque d'entraîner une baisse de la participation à la prise en charge des frais fixes spécifiques à la filière papier. Dans le contexte actuel d'explosion des coûts du service public de gestion des déchets, de la hausse future de la TGAP ou encore des coûts de l'énergie, les acteurs mettent en garde contre une nouvelle remise en cause des soutiens perçus par les collectivités pour les investissements qu'elles ont dû consentir afin d'améliorer, notamment, le tri spécifique des déchets de la filière papier.

part, les élus, notamment communaux, s'inquiètent du risque de déstabilisation de l'organisation des éco-organismes et de la future disparition de la filière papier, entraînant de nouvelles pertes. La fusion des deux filières soulève aussi des questions concernant le suivi des objectifs environnementaux : ils ne sont pas identiques de chaque côté et accusent déjà du retard. Est-il opportun de créer de l'incertitude en opérant cette fusion alors que de nouveaux objectifs ne sont pas clairement définis ? Le dernier point qui nous interroge concerne la faisabilité rapide de la fusion. Cette dernière devrait intervenir en 2024 avec, d'ici là, la publication d'un nouveau cahier des charges et le déploiement de la procédure d'agrément des acteurs autorisés à intervenir dans la nouvelle REP. Pour l'instant, seul l'un d'entre eux, en l'occurrence Citeo, bénéficie en 2023 de l'agrément pour les emballages ménagers et le papier. Concernant la prolongation de l'exemption de participation à la filière REP emballages ménagers et REP papier accordée à la presse, je rappelle que, depuis le 1 janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est soumise à une écocontribution. Comme tous les autres écocontributeurs, la presse devait ainsi participer au financement de la collecte, du tri et du recyclage. Compte tenu de la fragilité, invoquée ici et là, du modèle économique de la presse papier, il avait été décidé à l'époque que les éditeurs concernés pourraient bénéficier d'un régime spécifique. Ainsi, il leur serait possible de choisir de régler leur écocontribution en numéraire ou bien en nature, c'est-à-dire sous forme d'encarts publicitaires faisant la promotion de la transition écologique. Or la loi Agec tendait, à partir du 1 janvier 2023, à la suppression de ce régime particulier et à un alignement du mode d'écocontribution sur les autres secteurs.

par leurs activités. N'est-ce pas aussi un mauvais signal envoyé à diverses autres filières ? En effet, bien d'autres secteurs d'activité subissent la crise ; je pense notamment au BTP, dont l'activité est menacée par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Dès lors, chaque filière pourrait, à bon droit, demander un examen de sa situation particulière au regard de sa part de

Comme je l'ai indiqué lors de la discussion générale, je suis très attaché au maintien de la presse dans le champ de la filière REP. J'ai parfaitement conscience des difficultés de ce secteur, qui traverse une crise conjoncturelle et structurelle. Toutefois, je considère qu'il est impensable de remettre en cause le principe pollueur-payeur inhérent aux filières REP, dont l'importance est plus que jamais criante à l'heure de la crise environnementale que nous traversons et de la nécessité d'engager l'ensemble de notre système de production et de consommation dans la voie de la sobriété et de l'économie circulaire. À ce titre, tout le monde doit participer à l'effort collectif et aucun passe-droit ne doit être accordé. De plus, je reste convaincu qu'exempter un secteur du fait de ses difficultés économiques créerait un précédent ; beaucoup d'autres pourraient réclamer un traitement similaire, ce qui, à l'image du château de cartes qui s'écroule, mettrait à mal tout le système. Néanmoins, afin de tenir compte de la situation particulière de la presse, le présent amendement vise à maintenir l'autorisation des contributions en nature, sous la forme d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et sur le recyclage des papiers graphiques et autres déchets. Ce dispositif se matérialiserait sous la forme d'une convention signée et donc négociée par les trois parties prenantes, à savoir l'éco-organisme agréé, les collectivités territoriales et les entreprises concernées. C'est une solution de compromis

sur la forme, votre amendement n'est pas tout à fait compatible avec le droit européen. En effet, il a explicitement pour objet que la presse contribue en nature à la REP, ce qui n'est pas conforme à la directive Déchets de 2018, laquelle dispose que les metteurs sur le marché doivent contribuer financièrement à la filière à laquelle ils appartiennent. Toutefois, sur le fond, cet amendement est pleinement satisfait par la solution proposée par la commission, qui- je le rappelle -maintient la presse au sein de la REP et lui permet de bénéficier de primes en contrepartie de la mise à disposition d'encarts. Ces primes pourront conduire à l'annulation de sa contribution financière.

Nous proposons par cet amendement de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas d'exonérer la presse de toute responsabilité environnementale et de toute contribution à la prévention des déchets : cette dernière continuerait à s'appliquer en nature. Le système de modulation et de mutualisation introduit par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat demeure juridiquement fragile. Accorder une prime à la presse au titre de la REP en raison de la mise à disposition d'encarts ou du respect de certains critères de performance environnementale revient à maintenir une contribution en nature, en méconnaissance de la directive européenne du 30 mai 2018, qui a posé des exigences générales minimales applicables à la

La France est le seul pays européen à avoir instauré une REP sur les papiers graphiques, sans pour autant se révéler plus performante que d'autres pays qui ne l'ont pas instaurée. Un rapport d'information de l'Assemblée nationale publié en 2013 explique les raisons du faible taux de performance du recyclage en France et de son coût de traitement plus important

Il s'agit de prendre en compte les spécificités de ces deux filières ainsi que la différence importante de leur poids financier. En effet, l'écocontribution versée par les producteurs et distributeurs d'emballages ménagers serait de l'ordre de 900 millions d'euros par an, soit dix fois plus que l'écocontribution de la filière des papiers graphiques, qui varie entre 70 millions et 90 millions d'euros par an. La rapporteure a supprimé cette disposition en commission au motif qu'elle reviendrait à limiter les possibilités de synergie financière entre les emballages et les papiers graphiques, mais aussi au nom de la simplification. pour les sénateurs de notre groupe, il semble important, ne serait-ce que dans un premier temps, de maintenir cette différence pour s'assurer qu'aucune filière ne puisse pâtir de ce déséquilibre important et pour être certain, par là même, que le principe pollueur-payeur est bien respecté.

Si nous avons bien compris que ce n'est nullement l'objectif de la rapporteure, nous estimons néanmoins que renvoyer à un décret le soin de déterminer les conditions qui permettront de bénéficier de ces écomodulations fait courir un risque bien trop grand.

que ces critères comprennent l'écoconception, l'incorporation de matières recyclées et l'élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou la teneur en fibres recyclées.

par le texte de la commission, qui maintient la presse au sein de la REP et qui la fait bénéficier de primes en contrepartie de la mise à disposition d'encarts. Ces primes pourront conduire à l'annulation de sa contribution financière dès lors qu'elles seront valorisées à hauteur de l'écocontribution due.

Premièrement, votre proposition est juridiquement plus robuste que celle de la commission, dont les fragilités juridiques pourraient être contre-productives si le dispositif venait à être annulé. Nous nous retrouverions alors sans solution pour le secteur de la presse, alors même qu'il s'agit de notre préoccupation

que celui du Gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

sans prévoir en contrepartie un dispositif de compensation financière du manque à gagner qui en résultera pour la filière. Il décide par là même de se dédire, en revenant sur les dispositions de la loi Agec, qu'il a lui-même portée qu'il a lui-même portée et qui prévoyait la fin du régime dérogatoire de la presse écrite au 1janvier 2023. Madame la secrétaire d'État, nous partageons sur toutes nos travées des inquiétudes sur le devenir de la presse écrite. Pour autant, je le répète, exempter purement et simplement la presse de ses obligations n'est pas une solution pérenne. Cela créera un précédent : de nombreux secteurs également en difficulté demanderont sans doute un traitement similaire dans les prochaines années. Par ailleurs, cette exclusion représente un manque à gagner de l'ordre de 20 millions d'euros pour les collectivités territoriales, qui, elles, devront continuer à assurer la collecte, le tri et la gestion des déchets. Si le Gouvernement estime que les spécificités du secteur de la presse écrite justifient une telle exemption au principe général pollueur-payeur, il doit prendre ses responsabilités et prendre en charge le coût de cette décision, mais il ne doit en aucun cas le faire peser sur les autres contributeurs de la future filière REP fusionnée.

vous exposer. La réglementation en vigueur prévoit que les éco-organismes réalisent régulièrement une évaluation de l'impact des critères, des montants des modulations et de leur adéquation au regard des objectifs atteints. Par ailleurs, l'Agence de l'environnement

Les Républicains. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, pour conclure nos débats, je souhaitais, en ma qualité de président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, exprimer une double satisfaction et lancer un appel à nos collègues députés et au Gouvernement. Ma première satisfaction tient à l'esprit constructif dans lequel la commission a travaillé, pour soutenir Mme la rapporteure, qui s'est penchée pendant plusieurs semaines sur ce texte, aussi sensible, pour nos collectivités, que technique.